monsieur le président,

Cet amendement a pour objet d'attribuer un pouvoir général de prescription médicamenteuse aux médecins coordonnateurs des EHPAD. Je précise d'emblée que, en aucun cas,

doivent nécessairement faire intervenir le médecin traitant de chaque résidant, sauf urgence, bien entendu. Elle permettrait également de renforcer le rôle du médecin d'établissement, qui est bien souvent l'acteur médical principal et qui a, de fait, la plus grande proximité avec la personne accueillie.

madame la ministre,

à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles comme services médico-sociaux. Elles ont pour mission de veiller à l'accompagnement médical et social de personnes très démunies et atteintes de pathologies chroniques.

En outre, les établissements publics ont un EPRD unique, dès lors qu'un établissement social et médico-social est sous CPOM. L'EPRD permet de concilier transparence dans l'emploi des crédits et, surtout, souplesse de gestion accrue pour les organismes gestionnaires, afin notamment de pouvoir conduire la transformation de l'offre attendue par les pouvoirs publics.

a généralisé le système de l'EPRD pour les EHPAD, ce qui se traduit pour ces établissements par un assouplissement des procédures comptables, mais également un dialogue renforcé avec les autorités de gestion et de tarification. Par cet amendement, nous proposons d'étendre la possibilité d'adopter l'EPRD. Cette mesure pourrait simplifier la gestion comptable de ces établissements et les rapports avec les autorités. Elle représente aussi une mesure d'égalité entre établissements. Enfin, il s'agit d'une

visent à introduire une double mesure. En premier lieu, il s'agit de mettre fin à l'ingérence tarifaire en cours d'exercice de l'autorité de tarification et de contrôle pour tout établissement médico-social, et non plus et non plus seulement pour ceux dont les dotations sont préalablement définies par arrêté ministériel. En second lieu, il s'agit de préciser que tout établissement et service social et médico-social, à l'exception des EHPAD et des établissements accueillant des personnes handicapées, ne pourra se voir imposer le remplacement de documents budgétaires fondés sur une logique prévisionnelle par un état de prévision de recettes et de dépenses. La commission des affaires sociales est plutôt favorable à la première mesure, qui lui semble de nature à accroître la liberté gestionnaire, comme Elle est, en revanche, beaucoup plus réservée sur la seconde : la diffusion de l'EPRD et d'une logique budgétaire fondée sur un pilotage par l'activité semble être la contrepartie indispensable à la liberté gestionnaire. Par conséquent,

Cet amendement vise donc à supprimer l'obligation de transmission d'un budget primitif au 31 octobre pour les établissements publics. Afin de lever la contrainte de la double présentation budgétaire à laquelle sont confrontés les établissements publics relevant des dispositions de l'article L. 312-12-2 du code de l'action sociale et des familles, cet alignement est nécessaire.

mentionnés au IV de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles.

Un budget unique est évidemment plus lisible, et sa présentation au plus près de l'année à venir permet une projection plus fine que si elle intervient au début de l'automne. Le mécanisme actuel, associé à une réforme tarifaire

présentés par les directeurs d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux du cadre pluriannuel de la contractualisation, ce qui revient en droit à les rendre de nouveau dépendants d'une gestion strictement annuelle. Il me semble que cela ne va pas du tout dans le sens d'une plus grande liberté et efficacité gestionnaires. Par ailleurs, ils visent à exclure les EHPAD et les structures chargées de l'accompagnement des personnes handicapées de tout dialogue de gestion avec l'autorité tarifaire.

du Gouvernement ? Il est proposé de supprimer, pour les établissements publics qui ont signé un CEPOM et produisent un état prévisionnel des recettes et des dépenses, l'obligation de faire voter par leur conseil d'administration le budget prévisionnel avant le 30 octobre de l'année n-1. Tous les établissements publics ne sont pas contraints d'utiliser deux types de présentation budgétaire différents. Dès lors que l'établissement a signé un CEPOM, seul l'EPRD est à produire pour le 31 octobre. Par ailleurs, il nous semble souhaitable qu'un EPRD prévisionnel soit présenté au conseil d'administration avant le 31 octobre de l'année n-1. C'est un acte nécessaire, pour ne pas dire indispensable, pour la gestion de l'établissement et sa gouvernance que de voter le budget avant le début de l'exercice budgétaire. Par conséquent, le Gouvernement

pensé pour simplifier les obligations déclaratives des employeurs particuliers, est l'instrument tout désigné pour la rémunération par la personne accueillie de son accueillant. Il l'est néanmoins beaucoup moins pour assurer la couverture des frais professionnels, qui excède le champ de l'obligation déclarative ainsi que la compétence des URSSAF. Il n'en demeure pas moins que la rédaction de l'article visé par l'amendement prévoit déjà que le CESU puisse couvrir ces frais.

En effet, cette indemnité fait partie des contreparties financières prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, qui sont déjà visées par cet article. De plus, cette indemnité figure bien sur le bulletin de paie unique ou, plus exactement, sur le relevé de contreparties financières, qui est l'équivalent du bulletin de paie pour les accueillants familiaux et qui présente tous les éléments de la rémunération de l'accueillant. Cette demande étant déjà satisfaite, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

consiste, quand le tarif de soins d'un établissement excède un plafond national prédéfini, à le ramener au niveau de ce dernier. Afin de ramener les EHPAD au niveau des tarifs plafonds de soins fixés par la ministre de la sécurité sociale, est aujourd'hui proposée une mesure de réduction du délai de convergence tarifaire de sept ans Au regard des difficultés que rencontrent un certain nombre d'établissements, il nous semble indispensable de maintenir le délai de convergence initial pour les établissements en convergence négative, à savoir ceux dont les tarifs de soins sont au-dessus des tarifs plafonds, pour ne pas les pénaliser encore davantage. Quel commission ? Cet amendement vise à revenir sur l'accélération du rythme de la convergence tarifaire des EHPAD et à conserver le rythme actuel pour les établissements perdants sur le forfait soins. Il pose deux difficultés majeures. D'une part, il implique qu'un établissement pourrait perdre à la réforme tarifaire en cas de diminution de son forfait soins, alors que son équilibre budgétaire dépend également de son forfait dépendance. Par ailleurs, il ignore les efforts exceptionnels financés par le Gouvernement, qui, normalement, neutralisent totalement cet impact. D'autre part, il présente un risque manifeste d'inconstitutionnalité en introduisant une inégalité devant les charges publiques entre établissements.

En effet, certaines personnes ayant de réels besoins ne rentrent pas dans le périmètre défini par l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments

rénovation des prestations de compensation du handicap pour mieux prendre en compte les besoins des personnes. La problématique des aides techniques a été abordée dans le cadre de ce chantier, puisqu'elle a été explicitement évoquée lors du conseil interministériel du handicap. Nous avons d'ores et déjà engagé, en

ont mis en évidence une situation certainement sous-estimée et particulièrement préoccupante, aux conséquences très lourdes, d'abord bien sûr pour les patients, en termes de perte de chances et de confiance,

des efforts déployés par les entreprises pharmaceutiques pour garantir l'adaptabilité de leurs schémas de production aux variations de la demande et prévenir les risques de rupture de stock. notamment au doublonnage des sites de production ou à la mise en oeuvre de processus de fabrication innovants et plus réactifs, telle la fabrication en continu. Ces efforts requièrent des investissements qui devraient pouvoir être valorisés dans le cadre de la fixation du prix des médicaments par le CEPS. de la place de certaines spécialités anciennes dans l'arsenal thérapeutique particulièrement exposées à des risques de rupture de stock. Ces médicaments, qui s'adressent parfois à des populations cibles restreintes, font souvent l'objet d'une seule campagne de production par an en raison de leur faible prix. Je vous remercie

Vous souhaitez utiliser le prix comme un moyen de pression pour favoriser la production sur le territoire. Il ne nous semble pas que ce soit le bon moyen d'y arriver, d'abord parce que le prix n'est que très rarement une cause de

je souhaite vous faire part de notre perplexité, et même de notre inquiétude, devant la complexité de cet article. Cette complexité résulte pour partie de sa construction, puisqu'il recouvre plusieurs sujets n'ayant que peu à voir entre eux, depuis les extensions d'indication pour des médicaments de pointe jusqu'à l'évaluation de l'homéopathie, en passant par la régulation des médicaments en association. Il en résulte une intrication de dispositifs tout à fait illisible,

résulte également du fond des dispositions prévues : le degré de raffinement atteint par les divers dispositifs de prise en charge des produits de santé en rend la compréhension tout à fait inaccessible au profane, mais aussi aux sièges étrangers des grandes entreprises pharmaceutiques. Cette évolution me paraît contraire à l'esprit qui avait présidé

ne peut cependant que laisser pantois et desservir l'attractivité de la France pour les entreprises pharmaceutiques. Je souhaite maintenant relayer les inquiétudes exprimées par certains acteurs de santé que j'ai entendus au sujet du calendrier d'application des extensions d'indication. Il semble en effet qu'un certain flou entoure les potentielles

Comment ces extensions, qui concernent principalement les immunothérapies, semble-t-il, pourront-elles être rapidement mises à disposition des patients ? D'autres acteurs se sont émus de la formulation retenue dans l'article

Je n'approuve pas la proposition d'ouvrir le dispositif des autorisations temporaires d'utilisation aux extensions d'indication thérapeutique, d'autant qu'un précédent rapport sénatorial de 2011 préconisait, au contraire, de modifier le statut des ATU afin d'éviter que le titulaire des droits d'un médicament n'utilise cette voie à seule

constituait « une avancée majeure du projet de loi. L'ancien système donnait, en effet, lieu à un certain nombre de dérives : les autorisations temporaires d'utilisation étaient parfois utilisées par les laboratoires pour contourner l'autorisation de mise sur le marché, dans des conditions non encadrées et potentiellement dangereuses pour les patients. Or l'article 42 assouplit considérablement les règles du jeu. Actuellement, la procédure des extensions d'indication impose à l'industriel de déposer un nouveau dossier complet, qui doit être examiné par les différentes instances. Ce processus est donc nécessairement long, mais il me semble qu'il est aussi garant d'une certaine sécurité sanitaire. Il ne s'agit en

Mme la ministre.

sur l'article. Avec l'immunothérapie, on assiste à une révolution thérapeutique, un peu à l'instar de celle que l'on a connue il y a quelques dizaines d'années avec les antibiotiques.

les modalités autoritaires de fixation du prix par arrêté ministériel sont perçues comme un repoussoir et constituent un frein à la mise à disposition de ces traitements par les industriels. Afin d'assurer aux patients l'accès à ces innovations, il est proposé que les conditions économiques d'accès au marché soient négociées dans le cadre habituel de la politique conventionnelle, c'est-à-dire entre le comité économique des produits de santé et l'industriel. À défaut d'accord conventionnel, le ministère de la santé garderait la possibilité de décider du prix. Les mécanismes de régulation existants garantissent l'encadrement des dépenses de médicament. Cet amendement, du même ordre que le précédent, tend à prévoir, pour la détermination de la compensation applicable aux extensions d'indication et à l'accès direct en post-ATU, ainsi que pour le mécanisme d'accès précoce proposé pour les dispositifs médicaux, un mécanisme de négociation conventionnelle semblable à celui qui a communément cours en matière de fixation des prix des produits de santé.

ne jouera qu'en trésorerie, dans la mesure où le prix net négocié avec le CEPS viendra rétroactivement s'appliquer. Nous estimons cependant que le principe de la primauté conventionnelle doit continuer de régir l'organisation des soins comme la régulation des produits de santé. L'efficacité de l'action publique en matière de santé ne saurait découler que de la bonne implication et coopération de l'ensemble des acteurs concernés. En outre, dans un marché pharmaceutique mondialisé, le maintien de l'attractivité de la France constitue un enjeu majeur

notamment pour objet de prévoir que lorsqu'une spécialité pharmaceutique dispose d'une autorisation de mise sur le marché pour au moins l'une de ses indications et qu'une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l'article L. 162-16-5-1-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l'entreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de l'indication pour laquelle une prise en charge est autorisée.

pour laquelle une prise en charge est autorisée en application de cet article. Le présent amendement vise à garantir que la fixation de la compensation accordée en application des articles susvisés se fasse dans le respect des principes de la politique conventionnelle. Quel

Mme la rapporteur.

Une troisième approche repose sur le constat- je ne crois pas qu'il puisse être contesté -que la France est, parmi les grandes démocraties modernes, le pays où le médicament est le moins cher.

Delmont-Koropoulis. Le ministère des solidarités et de la santé a récemment demandé à la Haute Autorité de santé de mener une étude en vue d'évaluer l'efficacité des médicaments homéopathiques. L'homéopathie fait partie des pratiques courantes de soins de nos compatriotes. Un Français de soins de nos compatriotes. Un Français sur deux y a déjà eu recours. L'homéopathie a une véritable place dans la stratégie thérapeutique, et cela ne se limite pas aux maladies bégnines.

On constate, chez les patients pris en charge par un médecin homéopathe, une consommation deux fois moindre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et trois fois moindre de psychotropes. C'est également une alternative efficace et très employée à la prescription d'antibiotiques, notamment en pédiatrie. Dès lors, je demande que l'on m'explique quel serait l'intérêt économique d'un déremboursement des médicaments homéopathiques.

Outre son impact sur cette population, un arrêt arbitraire du remboursement de l'homéopathie serait une injure faite aux médecins homéopathes,

Eu égard à l'inscription des préparations homéopathiques à la pharmacopée française depuis 1965, au fait qu'un Français sur deux a déjà eu recours à l'homéopathie et à la faible part de celle-ci dans les dépenses de l'assurance maladie, il apparaît important de ne pas agir dans la précipitation, mais, au contraire, de privilégier la concertation pour la prise de toute décision concernant la prise en charge des médicaments homéopathiques par l'assurance maladie.

Le remboursement des médicaments homéopathiques représente 0,29 % des remboursements de médicaments par l'assurance maladie et 0,06 % de ses dépenses totales. Ces chiffres sont faibles. Néanmoins, en cas de déremboursement, les patients ayant recours à l'homéopathie risquent de se détourner de ces médicaments, au bénéfice d'autres, pris en charge par l'assurance maladie et plus coûteux. Cela aura pour effet pervers d'augmenter les dépenses de l'assurance maladie. Les médicaments homéopathiques sont une alternative thérapeutique aux soins classiques, encadrée par des professionnels de santé.

Sur le plan économique, la prise en charge des médicaments et préparations magistrales homéopathiques ne représente que 0,29 % des remboursements de médicaments supportés par l'assurance maladie et 0,06 % des dépenses totales. Si l'on mettait il y aurait inévitablement un report de prescriptions vers des médicaments plus chers et ayant davantage d'effets indésirables. Il est indispensable d'agir sereinement et de ne pas se limiter à écouter les oiseaux de mauvais augure. En effet, un Français sur deux a déjà eu recours à l'homéopathie et les traitements homéopathiques sont prescrits par un quart des médecins généralistes et par 78 % des sages-femmes, ou lors de consultations à l'hôpital, par exemple en oncologie. Ils sont disponibles dans

qui ne doit pas trop différer des méthodes d'évaluation des autres médicaments.

en accord avec les représentants des associations des homéopathes de France, afin de laisser le temps à cette concertation de s'organiser en toute sérénité et de porter ses fruits. Bien évidemment, je serai particulièrement attentive à son développement et à ses conclusions,

largement. Des obligations ont été instaurées l'an passé. Ces mesures de régulation apparaissent particulièrement ambitieuses pour un secteur économique en cours de structuration, qui repose encore principalement sur un réseau de petites entreprises produisant le plus souvent en petite série, avec un gain marginal faible. Par ailleurs, l'articulation avec la volonté de développer plus largement les prises en charge ambulatoires doit être clarifiée et, à cet égard, nous regrettons l'absence d'accord-cadre entre les entreprises du secteur et le CEPS. Dans l'attente d'une souhaitable remise à plat de la régulation financière des dispositifs médicaux, ces amendements tendent à modifier la liste des critères pouvant être pris en compte pour décider de la baisse du tarif de responsabilité de certains produits et prestations. Il s'agit tout d'abord- c'est l'objet de l'amendement n° 87 -de préciser que le critère du prix d'achat des produits et prestations

santé. La rédaction actuelle emporte une régulation strictement comptable, qui ne tient pas compte des besoins en santé de la population, ni des orientations par ailleurs décidées pour le développement de prises en charge non hospitalières. Quel est l'avis du Gouvernement

à Mme Laurence Cohen. Dans son rapport sur la fixation des prix des médicaments de 2017, la Cour des comptes a critiqué la mise à contribution de l'assurance maladie pour le financement de la politique industrielle des médicaments, alors que les entreprises bénéficient déjà d'une aide des pouvoirs publics au travers de la fixation du prix des médicaments, avec un crédit d'impôt recherche de 6,27 milliards d'euros. Si les entreprises qui exposent des dépenses de recherche et développement pour mettre au point de nouveaux traitements doivent effectivement intégrer ces coûts dans le prix du médicament,

dont l'amélioration du service médical rendu. Sont également pris en considération les résultats de l'évaluation médico-économique, le prix des médicaments à même visée thérapeutique, les volumes de ventes prévus ou constatés, ainsi que les conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Nous proposons de procéder à une évaluation la plus cohérente possible au regard des investissements effectifs, et de veiller à la soutenabilité du prix fixé pour le système de santé. Nous suggérons, dans cet esprit, de compléter la liste des critères pour la fixation des prix des médicaments prévue au code de la sécurité sociale et de permettre au Comité économique des produits de santé d'en tenir compte. Quel est l'avis de la commission ?

Dans son rapport de 2011, puis dans celui de 2017, relatifs à la sécurité sociale, la Cour des comptes alerte sur la faiblesse du cadre juridique de la révision des prix des médicaments. Elle déplore en effet que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ait précisé les critères de fixation des prix révisés, mais pas les cas de déclenchement de ladite révision. Nous proposons donc de clarifier le dispositif afin de combler ce vide juridique et de suivre ainsi les recommandations de la Cour des comptes, qui considère d'ailleurs que cette mesure permettrait à la sécurité sociale d'économiser des sommes considérables. Par exemple, en 2015, les économies liées aux baisses des prix des médicaments ont atteint 800 millions d'euros. On peut imaginer que ces économies seraient encore plus importantes avec des dispositions légales plus précises. Pour ces raisons, nous vous présentons cet amendement, qui prévoit trois cas dans lesquels le prix du médicament serait automatiquement révisé : à l'issue des cinq années de garantie de prix européen pour les médicaments les plus innovants ; à l'échéance de trois ans pour les autres médicaments ; en cas d'extension d'indication thérapeutique d'un médicament. Adopter cette mesure permettrait à la sécurité sociale d'économiser des sommes importantes et d'offrir un meilleur accès aux médicaments.

à l'article que vous souhaitez modifier, aux critères jusque-là utilisés par le CEPS pour déterminer le niveau du prix du médicament dans le cadre d'une procédure de révision. Dans la mesure où cet outil juridique est tout récent, il ne nous apparaît pas opportun de le modifier immédiatement

un avis défavorable pour trois raisons. D'abord, les critères de fixation des prix ont été révisés en 2017, et ils nous semblent pour l'heure suffisants. Ils permettent au CEPS de réviser les prix périodiquement, comme vous le souhaitez.

M. Philippe Mouiller. La régulation des dépenses de santé est un enjeu majeur, qui doit être corrélé aux ambitions sous-tendant la stratégie nationale de santé et le plan Ma santé 2022, qui visent notamment à garantir et à promouvoir la pertinence des soins. En conséquence, c'est au regard de ce critère que doit être apprécié le bien-fondé des dépenses de santé, et non sur la base de mécanismes de baisse uniquement comptables des dépenses, sans lien avec les besoins médicaux et la pertinence de soins.

Je suis, par ailleurs, d'accord avec M. Mouiller sur le fait que le mode de régulation des dépenses de produits de santé est à revoir, en raison principalement de sa trop grande complexité. Selon nous, cette régulation doit prioritairement passer par la voie conventionnelle. Une refonte de l'accord-cadre entre le CEPS et les entreprises du médicament et la mise en place d'un accord-cadre pour les dispositifs médicaux

à plus de quinze ans, notamment dans le traitement des troubles neurodégénératifs, dont l'évolution est très lente. Ces lenteurs induisent des pertes de chances pour les patients et mettent en danger des sociétés de biotechnologies innovantes, qui se retrouvent à court de financements, et ce même après l'obtention de résultats prometteurs. La mise à disposition de médicaments contenant certaines molécules ayant démontré leur potentiel thérapeutique se trouve freinée par le cadre juridique actuel applicable aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, mais également aux demandes d'ATU, au-delà des incontournables difficultés associées à la prise en charge par l'assurance maladie de ces modes d'accès aux médicaments. Si certaines autorisations temporaires d'utilisation peuvent être octroyées à un stade assez précoce de développement, elles sont, par définition, subordonnées à une autorisation délivrée par l'autorité compétente sur la base de la démonstration tant de la sécurité que de l'efficacité d'emploi du médicament concerné. Or certains patients faisant face à une maladie incurable souhaitent pouvoir bénéficier de ces médicaments innovants en prenant, de manière éclairée, de manière éclairée, et donc en toute connaissance de cause, le risque thérapeutique associé à leur utilisation. Ce droit à la recherche de leur survie doit leur être reconnu et garanti. L'introduction de ce dispositif, qui serait un nouveau mode légal d'accès aux médicaments, au côté de l'AMM et de l'ATU, permettrait de réduire dans des proportions considérables les délais imposés

neuroprotectrices présentent par nature un profil de sécurité encourageant. Le financement de cette voie d'accès nouvelle serait en partie assuré par un fonds de solidarité constitué par une participation des laboratoires ayant recours au dispositif de l'UTES.

Cet article, qui a été inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation de l'ouverture des ATU aux extensions d'indication dans les deux années suivant la promulgation de la loi. Le sujet du rapport proposé ne manque pas d'intérêt, car le suivi des extensions d'indication prises en charge dans le cadre des ATU devra faire l'objet d'une attention particulière.

Si nous sommes conscients de l'importance de développer le recours aux médicaments génériques pour alléger les comptes de la sécurité sociale, cela ne saurait s'accomplir au détriment de la santé de nos concitoyens. Or cet article crée une nouvelle catégorie de médicaments, les hybrides, que le pharmacien pourra substituer aux médicaments originaux. Les médicaments hybrides, à peine connus du grand public, sont fabriqués à partir des mêmes principes actifs que le médicament principal, mais selon des posologies, sous des formes ou pour des indications complètement différentes. Nous ne disposons pas du recul nécessaire et de garanties sanitaires suffisantes pour généraliser l'usage de ces nouveaux médicaments. et Territoires est donc fermement opposé à cette mesure. Nous invitons le Gouvernement à la plus grande prudence, dans l'intérêt de tous. Nous considérons également que le médecin doit rester maître de la décision de remplacer ou non un médicament par un générique et, à plus forte raison, par un hybride.

La notion de médicament hybride est en effet largement absente du débat public et n'a pas fait l'objet de travaux ni de conclusions particulières dans le cadre du

L'interchangeabilité des produits inhalés pose encore de nombreuses questions en matière de sécurité sanitaire, notamment liées à la nécessité d'une éducation thérapeutique des patients, compte tenu de la variabilité des mécanismes d'utilisation par voie inhalée.

: La parole est à M. Fabien Gay. Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 22 à 33 de cet article, qui introduisent la possibilité de limiter les remboursements de médicaments au tarif en vigueur pour les médicaments génériques ou hybrides. Autrement dit, ces dispositions limitent le remboursement des médicaments princeps. Présentées comme une incitation à consommer prioritairement des médicaments génériques, elles constituent en réalité une sanction contre les patients. Nous rappelons que ceux-ci disposent d'une liberté de choix thérapeutique, qui doit leur permettre de choisir non seulement les actes qu'ils subissent, mais également les traitements qui leur sont administrés. La réduction des remboursements pour les traitements princeps vient porter atteinte à cette liberté. Certes, cette disposition n'interdit pas explicitement le recours aux médicaments princeps, et une personne qui ne souhaite pas avoir recours aux génériques pourra toujours acheter le médicament de son choix en pharmacie. Mais ce dispositif vient limiter la liberté de choix des usagers du service public de la santé les moins aisés.

vise à supprimer la prise en charge par l'assuré de la différence de prix entre le princeps et le générique le plus cher. Pour notre part, nous proposons une stratégie concertée entre médecins et pharmaciens pour le développement des génériques.

amendement vise tout d'abord à supprimer la restriction du recours par les prescripteurs à la mention « non substituable ». Suscitant l'opposition de l'ensemble des acteurs concernés, cette mesure paraît en effet devoir rester inopérante en pratique, voire contre-productive.

encadrant les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, les CAQES. Ces contrats visent le même objectif d'amélioration de la pertinence du recours aux produits de santé.

En 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament a reçu 530 signalements de traitements « essentiels » en rupture de stock ou en tension d'approvisionnement. C'est du jamais-vu. Le nombre des cas de signalement de médicaments en tension d'approvisionnement ou en rupture de stock a été multiplié par plus de dix en moins de dix ans. Notre pays- dois-je le rappeler ? -est tout de même la septième puissance économique mondiale. Dès lors, comment accepter que ces pénuries surviennent et remettent en cause les traitements des patients, la continuité de leurs soins ? C'est ce constat qui a incité la commission des affaires sociales à se pencher sur la question et à mener un travail approfondi dans le cadre d'une mission d'information.

Il s'agit de créer une cellule nationale de gestion des ruptures d'approvisionnement, placée sous l'autorité du Premier ministre et chargée de définir une stratégie nationale pour la prévention et la résolution des causes de rupture d'approvisionnement. permettrait de renforcer la coordination dans la prévention et la gestion des tensions et ruptures d'approvisionnement. Quel

Avec cet amendement et celui que je présenterai ensuite à l'article 44, notre commission entend prendre part au débat contradictoire sur la réforme des retraites que souhaite le haut-commissaire

le niveau de vie des retraités. Toutes les expériences étrangères de réforme systémique le montrent, la question de l'âge minimum légal, au-delà de l'âge pivot, est centrale. Même les Suédois réfléchissent à relever cet âge minimum, pour protéger les femmes et les travailleurs les moins qualifiés contre le risque de partir trop tôt, avec une retraite insuffisante. À nos yeux,

Nous avons également indiqué que les Français se trouvant à moins de cinq ans de l'âge du départ à la retraite lors de l'adoption de la réforme ne seraient pas concernés. Or vous proposez de modifier un paramètre fondamental en 2020.

Dans le contexte actuel de réforme de l'ensemble du système, cette proposition fait figure à la fois de chiffon rouge et de leurre. Seule la réforme d'ensemble à laquelle travaillent

En effet, pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, le recours au temps partiel s'accentue avec l'âge. Les 55-64 ans ont 1,5 fois plus de chances de travailler à temps partiel que les 30-54 ans et 2 fois plus de chances que ce soit pour des raisons de santé.

en baisse de 1,3 % pour les plus de 55 ans et de 1,2 % pour les 60-64 ans. En France, une forte proportion des chômeurs de longue durée ont plus de 55 ans. Mes chers collègues, ces réalités m'interdisent de voter cet amendement ; je le dis au nom de la justice et de la cohésion de notre société.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

Ce dispositif déroge totalement à la règle selon laquelle les prestations sont revalorisées annuellement au niveau de l'inflation constatée sur l'année précédente, qui est de l'ordre de 1,6 % à 1,7 %.

selon lequel s'est bâtie notre protection sociale depuis des décennies. Il a permis jusqu'à maintenant de garantir le pouvoir d'achat de nos concitoyens, en particulier des plus modestes d'entre eux. Vous vous attaquez aux prestations familiales, aux pensions de retraite, aux pensions d'invalidité, aux rentes accident du travail-maladie professionnelle ou encore aux aides au logement : rien de moins ! Pour les retraités, cette décision intervient alors que l'année 2018

Ajustement exceptionnel », « revalorisation maîtrisée », « désindexation », « revalorisation différenciée », « sous-indexation » : on nous noie sous des formules complexes, en martelant qu'il y aura des gagnants. Pour ma part, je vois surtout des perdants Que l'on ne nous parle plus de gains de pouvoir d'achat, c'est exactement l'inverse ! Pour toutes ces raisons, nous présenterons un amendement visant à supprimer cet article profondément injuste et inégalitaire.

Après la hausse de la CSG, qui concerne plus de 7 millions de retraités, l'absence de toute revalorisation des pensions en 2018, impliquant une baisse de leur pouvoir d'achat, les retraités pouvaient espérer que leurs pensions seraient

Rappelons enfin que M. Delevoye, le haut-commissaire nommé par le Président de la République, préconise l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. La position du Gouvernement est simple quand l'inflation réapparaît, la désindexation des prestations sociales devient un outil très efficace de régulation des dépenses publiques. L'étude d'impact le prouve : en 2019, cette revalorisation permettra d'économiser 3,5 milliards d'euros ; en 2020, le gain sera proche de 7 milliards d'euros. Madame la ministre, mes chers collègues, le retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale doit être mis au service de la modernisation de notre système de santé et du progrès social. L'enjeu,

de dire la vérité aux gens. Nous aurions pu, comme le gouvernement précédent, proposer une augmentation de la durée de cotisation,

Nous avons fait le choix d'une revalorisation différenciée des prestations et d'un effort spécifique à destination des Français les plus modestes.

Aujourd'hui, nous revalorisons l'aide à la garde d'enfant pour les familles dont un enfant est handicapé et nous allongeons le congé de paternité.

la politique que je mène sont tournés vers les retraités les plus modestes ! Enfin, nous menons une politique ambitieuse de transformation de notre modèle de prise en charge des personnes âgées, avec

Il en va de même pour les familles, qui ont participé ces cinq dernières années à l'effort de modération des dépenses sociales. Le groupe Les Indépendants avait souhaité, dans un premier temps, limiter cette perte de pouvoir d'achat, tout en respectant l'exigence de préservation de l'équilibre des comptes sociaux. Tel était l'objet de l'amendement n° 226 rectifié de Daniel Chasseing. En définitive, nous nous rangeons aux arguments de la commission

qui est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l'allocataire est supérieur à 39 000 euros en France hexagonale et à 100 000 euros dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

de la commission ? Il est proposé d'expérimenter dans les outre-mer l'exclusion de la résidence principale de l'assiette de récupération sur succession de l'ASPA.

? Je ne répèterai pas ce que vient de dire M. le rapporteur. Je rappellerai simplement que la récupération sur succession est la contrepartie du fait que l'allocation du minimum vieillesse se substitue à l'obligation de solidarité

possèdent un petit héritage familial, un lopin de terre. Je pense principalement à toutes les communes de La Réunion, mais aussi de Guadeloupe et de Martinique,

Nous avions déposé un amendement sur cet article, mais il est tombé sous le couperet de l'article 40, ce qui ne me permettra pas de vous le présenter. Je souhaitais juste avoir, madame la ministre, votre avis sur un point, maintenant ou à un autre moment.

Pourtant, la loi de 2005 établit un lien direct entre l'attribution d'une pension d'invalidité et la reconnaissance d'un handicap. Pourquoi ne pouvons-nous pas considérer ces deux situations familiales sous le même prisme, pour plus d'équité et de transparence ?

du mode de garde, pour les familles dont l'enfant n'a pu être accueilli en école maternelle jusqu'à la rentrée scolaire suivant son troisième anniversaire. Si ces mesures vont dans le bon sens, elles suscitent une inquiétude grandissante dans certains territoires,

contre moins de 70 % en Guyane et à Mayotte. Il est vrai que le taux de scolarisation remonte ensuite fortement : il est d'environ 94 % pour les enfants âgés de quatre à cinq ans, ce qui peut se comprendre. Mais compte tenu des difficultés rencontrées dans ces académies à chaque rentrée scolaire, l'abaissement à trois ans pose mécaniquement un défi immense, tant en termes d'infrastructures que de ressources humaines. Rappelons que Mayotte est le seul territoire de la République où la double vacation existe.

ans et plus, puis j'y ai renoncé. Je me suis ensuite rappelé, avec regret, que ce même CMG n'était pas encore applicable à Mayotte, en dépit du plan « Mayotte 2025 », qui prévoit justement de favoriser la garde d'enfants. Enfin, il eut été finalement trop défaitiste de proposer un tel amendement, car je veux croire que nous serons en mesure d'accueillir tous ces enfants dans nos écoles à la prochaine rentrée. J'ai récemment interpellé à ce sujet le ministre Jean-Michel Blanquer, qui m'a assuré de son volontarisme.

Il ne faudrait pas que les familles soient doublement pénalisées : que leurs enfants ne soient pas scolarisés et qu'elles ne puissent bénéficier du CMG à taux plein. Mme Viviane Malet. Cet amendement vise à conserver la logique actuelle du versement de l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, dès le début de la scolarité obligatoire, sous condition de ressources, afin que les familles continuent à être aidées lors de la rentrée scolaire. La scolarisation des enfants entraîne des frais que certaines familles peuvent avoir des difficultés à prendre en charge, et ce dès l'école maternelle. Je pense notamment aux frais d'assurance, de cantine, de déplacement, de garderie

trois ans dès la rentrée 2019. Cette mesure purement comptable est en totale contradiction avec le plan de lutte contre la pauvreté. Nous le déplorons. l'ARS et l'âge de la scolarité obligatoire doivent donc être couplés sur la même base. Néanmoins, parce que nous sommes réalistes, nous prenons en considération le fait que les dépenses liées à l'entrée en maternelle sont inférieures à celles qui résultent de l'entrée en primaire. Par conséquent, le décret fixant le montant de l'ARS doit considérer une nouvelle tranche d'âge de trois à six ans, pour laquelle le montant de ladite allocation sera inférieur à celui qui est prévu pour les enfants de plus de six ans.

Cohen, sur l'article. L'article 47 prévoit d'harmoniser les modalités d'indemnisation du congé maternité, en particulier pour les travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles, avec celles du régime plus avantageux des salariées. Le projet de loi prévoit d'aligner la durée minimale d'arrêt pour les travailleuses indépendantes sur celle des salariées, soit huit semaines, dont deux de congé prénatal. En outre, la durée de versement maximale des indemnités journalières sera portée par décret à 112 jours, comme pour les salariées. Cet article va globalement dans le bon sens et tente de répondre à un problème que nous avions déjà soulevé,

allons prendre est évidemment importante, car il ne faudrait pas que la mesure proposée induise des effets pervers et conduise ces femmes à renoncer à des indemnités. À l'inverse, il ne faudrait pas que la souplesse introduite par le Sénat soit perçue comme un renoncement à accorder à ces femmes un droit supplémentaire.

européenne sur le congé maternité. Pour rappel, le texte prévoit d'allonger de quatorze à vingt semaines la durée minimale du congé maternité dans l'Union européenne. Les dispositions prévues par par cette directive permettent des avancées concrètes en faveur de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Cette directive est déterminante pour garantir l'autonomie économique des femmes, leur égal accès au marché du travail et un autre partage des tâches, sachant que la maternité et la parentalité sont parmi les premiers facteurs discriminants dont souffrent les femmes. En conclusion, le

de porter à huit semaines la durée minimale d'arrêt pour les travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles, dont deux semaines de congé prénatal, à l'instar de la durée appliquée aux salariées, pour bénéficier d'une indemnisation de leur congé maternité. Améliorant l'attractivité du dispositif, cet article prévoit également de supprimer le versement de la CSG et de la CRDS par les exploitantes agricoles bénéficiant de l'allocation de remplacement. L'article prévoit ensuite l'instauration d'une indemnité journalière forfaitaire en cas de maternité ou d'adoption. Cette indemnité strictement subsidiaire, accordée uniquement dans les cas où l'allocation de remplacement ne peut être versée, constituera un revenu de remplacement au même titre que pour les salariées et les travailleuses indépendantes non agricoles. de ces dispositions est de permettre à l'ensemble des femmes, en France, de bénéficier d'un congé maternité complet et effectif. En ce sens, cet article répond à l'engagement du Président de la République de réformer le congé maternité.

entre travailleuses de professions et de statuts différents, certes, mais bel et bien toutes confrontées à la nécessité de concilier contraintes professionnelles et impératifs familiaux. Cet amendement vise à mieux protéger les travailleuses indépendantes pendant leur congé maternité, en revenant sur la mesure proposée par le Gouvernement, qui conditionne le bénéfice des prestations de maternité pour ces travailleuses à une durée minimale d'interruption d'activité de huit semaines. Cette formulation peut apparaître paradoxale. Le dispositif que vous défendez, madame la ministre, est présenté comme étant plus protecteur de ces travailleuses, en ce qu'il aligne la durée minimale de leur congé maternité sur celle du congé des salariés. Il répond donc en théorie à un objectif de santé publique et d'harmonisation des droits que je ne puis que saluer. Je crains toutefois que, en pratique, il ne conduise certaines de ces travailleuses à se trouver contraintes de renoncer à toute forme d'indemnisation. Les conditions d'activité des travailleuses non salariées ne sont pas comparables, en effet, à celles des salariées. Certaines doivent assurer une activité dans les semaines qui précèdent leur accouchement pour garantir la viabilité de leur entreprise. Leur situation n'est donc pas comparable à celle des salariées, qui retrouvent leur poste à l'issue de leur congé. Je pense donc que la mesure proposée pourrait se révéler désincitative. Elle pourrait conduire certaines femmes à privilégier la poursuite de leur activité plutôt que le bénéfice des prestations de maternité afin de sauvegarder leur outil de travail pour l'avenir. Il pourrait au total en résulter une dégradation de l'indemnisation du congé de maternité pour ces travailleuses, à rebours de l'objectif affiché. En l'état actuel du droit, elles bénéficient d'une allocation de repos maternel d'un montant de 3 300 euros, sans condition d'interruption d'activité, et d'indemnités journalières de 54 euros par jour, à condition de s'arrêter au au moins 44 jours. Désormais, celles qui s'arrêteront moins de 56 jours n'auront plus droit à rien. Je considère que c'est un recul de leurs droits. En d'autres termes, si l'alignement l'alignement de la durée maximale de versement des prestations apparaît tout à fait souhaitable et plus protecteur, il n'en va pas de même s'agissant de la durée minimale d'interruption d'activité conditionnant le versement des prestations. Au regard de ces observations, et pour rester dans le cadre fixé par l'article 40 de la Constitution, l'amendement de la commission vise à régler les situations des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles de manière différenciée. Pour les travailleuses indépendantes, il est proposé de revenir au droit existant, plus protecteur en ce qu'il ne conditionne pas le versement des prestations à une durée minimale d'interruption d'activité. Pour les exploitantes agricoles, pour lesquelles le présent article comprend par ailleurs des avancées, nous proposons de renvoyer la définition de la durée minimale de cessation d'activité à la voie réglementaire. Afin de ne pas pénaliser les femmes qui pourraient se trouver contraintes de reprendre leur activité rapidement pour garantir la pérennité pérennité de leur entreprise, j'estime que cette durée minimale devrait être plus proche de trois à quatre semaines. Quel

En effet, le Gouvernement a souhaité, afin de préserver la santé des mères et des enfants, les inciter à prendre un véritable congé maternité et à renforcer leurs droits, selon les préconisations du rapport de Mme Marie-Pierre Rixain sur le congé de maternité, lequel a fait l'objet d'une large concertation. Les préconisations étaient, d'une part, d'aligner la durée globale du congé maternité sur celle dont bénéficient les salariées de 74 à 112 jours, et, d'autre part, d'augmenter la durée minimale d'interruption obligatoire de l'activité de 44 à 56 jours, soit 12 jours de plus,

de concilier congé maternité et reprise d'activité. Après l'arrêt obligatoire de huit semaines, les travailleuses indépendantes ont la possibilité de reprendre leur activité à temps partiel. contraire, conduirait les travailleuses indépendantes à renoncer à tout ou partie de leur congé, au détriment parfois de leur santé et de celle des enfants, plutôt qu'à essayer de l'aménager. C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut,

attendent une meilleure adéquation de la législation à leur activité professionnelle. Ce sont des spécificités de lisibilité, de flexibilité, de souplesse, de préservation de leur outil de travail. Ces besoins

L'article 47 prévoit d'aligner la durée minimale d'interruption d'activité ouvrant droit à des prestations de maternité pour les travailleuses indépendantes sur celles des salariées. Si cette mesure part d'un bon sentiment, elle risque d'augmenter le non-recours au droit au congé de maternité par ces femmes, sur lesquelles repose le fonctionnement de leur entreprise. Nous souhaitons que toutes les femmes puissent accéder de la même manière à l'interruption d'activité lors d'une maternité,

où le médecin n'est pas toujours accessible. Elle placerait en plus la sage-femme dans un cadre de coordination des soins entre praticiens, conformément à l'un des objectifs de ce PLFSS. En 2011, le rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale recommandait déjà de mieux articuler et de valoriser les compétences des sages-femmes, en faisant d'elles encore davantage des professionnelles de premier recours pour le suivi des femmes en bonne santé. Cette mesure constituera de plus une source d'économies pour la sécurité sociale, dès lors que les femmes enceintes ne seront plus tenues, comme c'est le cas aujourd'hui, de consulter leur médecin traitant pour obtenir la prescription d'examens que les sages-femmes sont déjà en mesure de prescrire. De fait, cela éviterait une double consultation. Quel est l'avis de la commission ? Avis favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

et leur champ d'intervention auprès des patientes. Je rappelle d'ailleurs que ce champ d'intervention a été élargi dans le cadre de l'avenant n° 4 de la convention nationale signée le 29 mai dernier entre les sages-femmes et l'assurance maladie. Cet avenant maintient et renforce la participation des sages-femmes à la mise en oeuvre des priorités de santé publique

-en permettant de récupérer des indus de prestations sur tous les autres, sans distinction, y compris les minima sociaux et les prestations en espèces de l'assurance maladie. Les dispositions de cet article feraient peser sur les personnes fragiles économiquement la mauvaise gestion des administrations.

de cet amendement, réduire le budget alloué aux soins de ville et répartir l'excédent en direction des cinq autres pôles de dépenses, notamment les établissements de santé, les établissements et services pour personnes âgées

EHPAD. La construction de l'ONDAM doit se fonder sur la réalité des parcours de soins des patients et traduire des priorités de santé publique. Tel qu'il est construit aujourd'hui,

2018 va constituer le sixième exercice excédentaire consécutif pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, AT-MP. Celle-ci a apuré l'intégralité de sa dette en 2016, de sorte que son solde cumulé pourrait avoisiner les 5 milliards d'euros en 2020. Les voyants sont au vert, ce qui ne signifie pas que les choses doivent rester en l'état. En effet, il convient, tout d'abord, d'accroître les actions de prévention, qui représentent aujourd'hui moins de 3 % des dépenses de la branche, mais aussi d'adapter cette dernière à son époque, en reconnaissant de nouveaux risques professionnels. Je pense au premier chef au fléau de l'épuisement professionnel, plus connu sous le vocable de burn-out. Ce dernier prend de l'ampleur. Le barème indicatif des maladies professionnelles ne correspond plus à la réalité des pathologies psychiques liées à la souffrance au travail. Son inadaptation empêche, de fait, toute reconnaissance réelle de ces dernières. Je souhaite donc que la concertation lancée par le Gouvernement sur la question de la santé au travail permette de formuler des propositions sur ces pathologies connues, qui ne peuvent demeurer non reconnues. Outre cette problématique du burn-out, je regrette que le Gouvernement n'ait pas profité de l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales avec le secteur agricole et alimentaire pour mettre en place un fonds d'indemnisation

Les malades, victimes de pathologies professionnelles ou environnementales, n'ont plus le temps d'attendre. Il faut agir, c'est une question de justice sociale ! Un amendement sera déposé sur ce sujet, et un autre visera le chlordécone, pesticide reconnu comme cancérogène et perturbateur endocrinien, utilisé durant plus de vingt ans dans les bananeraies et qui a pollué pour des siècles des écosystèmes antillais. Le fonds d'indemnisation que nous voulons créer a le mérite d'indemniser intégralement les victimes et d'être financé selon le principe du pollueur-payeur. Ce qui a été fait pour l'amiante doit être élargi. Nos concitoyens, partout en France, attendent que nous avancions sur ces questions.

dans le rapport remis au Premier ministre sur la santé au travail, socle de la concertation en cours- je l'évoquais tout à l'heure. Il nous apparaît nécessaire que le projet de loi vise également une amélioration du système d'indemnisation des maladies professionnelles pour les victimes du travail. Nous pensons en particulier à une meilleure reconnaissance des troubles psychosociaux et du syndrome d'épuisement au travail, qui font partie des maladies hors tableau et que la condition du taux d'incapacité de 25 % empêche aujourd'hui de reconnaître comme maladies professionnelles en tant que telles.

Le rapport de la commission d'évaluation de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles se penche d'ores et déjà sur la problématique des pathologies psychiques liées au travail, qui font l'objet d'une voie dérogatoire pour leur reconnaissance comme maladie professionnelle au travers des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

l'échelon national, cette approche maximaliste de certaines CARSAT soulève des difficultés, que ce soit un problème d'équité entre les maîtres d'ouvrage, une incohérence patente entre les différents codes de la construction et de l'habitation, du travail et de la sécurité sociale, qui place les maîtres d'ouvrage dans l'insécurité juridique, juridique, ou un impact financier souvent non négligeables des surprescriptions, qui se traduit par des travaux ou cotisations supplémentaires en cas d'inobservation de la recommandation des CARSAT. Au regard des lourdes conséquences juridiques et économiques pour les entreprises, cet amendement tend à préciser que, lorsque la loi ou le règlement prévoit des mesures alternatives, une CARSAT ne saurait « inviter » un employeur à recourir obligatoirement à l'une de ces mesures ou, inversement, à exclure l'une de ces mesures. Il consacre également la faculté des CARSAT de faire monter à l'échelon national une faille des mesures de prévention qu'elles auraient pu identifier, afin de permettre au pouvoir réglementaire d'harmoniser les mesures de prévention sur l'ensemble du territoire. Quel est l'avis de la commission ? En tant

Dans la prévention de certains accidents du travail présentant un fort risque de mortalité, il est parfaitement légitime que les CARSAT proposent des mesures complémentaires adaptées au contexte particulier de chaque entreprise. Il y va de la sécurité des salariés, et il revient

donc, à travers cet amendement, d'inscrire un rendez-vous régulier d'évaluation, et donc d'évolution potentielle des tableaux de maladies professionnelles, sur le fondement d'une expertise scientifique. L'amendement

par décret les tableaux de maladies professionnelles. L'évolution législative que nous proposons nous semble nécessaire, mais l'État aura la responsabilité de s'emparer de ces points d'étape triennaux pour acter les modifications nécessaires, dans l'intérêt des personnes concernées. Je voudrais enfin remercier

que nous avons reçue de la part de victimes de l'amiante. En effet, il est toujours complexe de faire reconnaître son exposition à une matière dont on sait pourtant qu'elle a tué, et qu'elle continue de tuer, des centaines de milliers de personnes dans le monde, notamment en France. Qu'il s'agisse de faire valoir ses droits de victimes ou de faire reconnaître un site comme amianté, c'est toujours un parcours du combattant, doublé d'une course contre la montre. Ma collègue Cathy Apourceau-Poly a d'ailleurs été interpellée récemment par des agents de la SNCF qui souhaitaient faire reconnaître la présence d'amiante dans les ateliers, qui sont bloqués par la raison d'État. En effet, reconnaître l'exposition à l'amiante de quelques cheminots, c'est reconnaître tous les ateliers comme potentiellement amiantés, avec le risque de sommes importantes à débourser par l'État. Nous sommes ici dans le cas plus précis de travailleurs souhaitant faire valoir leur droit à l'allocation pour cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'ACAATA, et qui se trouvent en contradiction, voire en opposition avec certaines CARSAT. En effet, il semblerait que certaines d'entre elles ne tiennent pas compte de la correction effectuée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et opposent une fin de non-recevoir aux potentiels allocataires, dès lors que ceux-ci auraient été exposés alors qu'ils étaient affiliés à un régime spécial. C'est particulièrement vrai pour les marins et dockers à Calais, Dunkerque ou ailleurs, qui ont été exposés des années durant à la fibre d'amiante et qui ont des difficultés à percevoir cette allocation. Par cet amendement de réécriture, nous souhaitons assurer une base légale claire au respect des droits de ces travailleurs. Quel

que ceux qui avaient relevé d'un seul régime. La rédaction actuelle de cet article permet donc déjà le cumul des périodes travaillées dans les établissements où le salarié a été exposé à l'amiante, que l'intéressé soit affilié au régime général ou à un régime spécial.

l'avis de la commission ? Le Président de la République s'est engagé, à la fin du mois de septembre 2018, à la reconnaissance comme maladie professionnelle de l'exposition au chlordécone.

? Madame la sénatrice, nous avons tenu les engagements que nous avons pris, puisque les travaux visant à la création de tableaux de maladies professionnelles ont été lancés par les instances dédiées de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et du régime agricole. Ces deux instances, composées des administrations concernées, des partenaires sociaux et des organismes d'expertise, ont inscrit la thématique des produits phytosanitaires, dont le chlordécone, dans le programme de travail pour de définir quelles seront les maladies reconnues pour les travailleurs exposés. Ces instances s'appuieront sur l'expertise scientifique de l'INSERM, qui a été saisi

Il tend à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits. à restreindre le champ de son action aux maladies d'origine professionnelle. Son adoption répondra ainsi à certaines inquiétudes et permettra l'adoption de ce dispositif majeur.

rapport n'a pas été rendu. Je rappelle que, parallèlement, nous avons demandé une expertise collective à l'INSERM et à l'ANSES pour bien définir les maladies

sur les cotisations des employeurs. Ce dispositif consisterait à augmenter les taux de cotisation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, lorsque les entreprises présentent une sinistralité anormalement élevée par rapport aux autres entreprises exerçant des activités similaires. Cette mesure a un double objectif. Le premier est d'inciter les entreprises à avoir de bonnes pratiques en termes de sécurité et de sanctionner les employeurs qui n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques. En effet, la loi impose aux employeurs une obligation de sécurité à l'égard de leurs salariés et, si un employeur manque à son obligation, il est légitime qu'il soit sanctionné, d'autant que ce manquement a des répercussions directes sur les salariés. Le second

En effet, il s'agit d'une sorte de forfait, qui ne tient pas réellement compte de la situation de l'entreprise ou de sa taille, traitant de la même façon par exemple une petite association et une grande entreprise. Le dispositif que nous vous proposons est plus juste, car il est fondé sur les cotisations sociales. Il prend donc en compte la taille de l'entreprise et le nombre de ses salariés. Quel est l'avis de la commission ?

À partir de 2022, le dispositif « prime-signal » permettra par exemple de majorer le taux de cotisation des entreprises de 10 à 19 salariés ayant des accidents du travail récurrents, dans la limite de 10 %. Par ailleurs, le code de la sécurité sociale autorise déjà les CARSAT à appliquer une cotisation supplémentaire aux entreprises qui méconnaissent leurs obligations en matière de prévention. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

à créer à cet effet une commission, présidée par un magistrat de la Cour des comptes, chargée de rédiger et publier ce rapport le 1 janvier de chaque année. L'Observatoire des non-recours aux droits et services, l'ODENORE, a dressé la typologie du phénomène de non-recours aux minimas sociaux, mais aujourd'hui nous sommes dans l'incapacité de chiffrer ce taux de non-recours. Or, afin de lutter contre ce fléau, il est incontournable de disposer d'une information précise et détaillée sur le sujet. Une prestation sociale est accessible, si elle trouve son public et si la fraction de la population qu'elle est destinée à aider la reçoit. Sinon, son service social rendu est faible, son utilité aussi. La persistance d'un taux de non-recours élevé à une prestation doit inciter les pouvoirs publics à réexaminer la façon même dont elle a été conçue

La lutte contre le non-recours aux droits est l'un des objectifs majeurs de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Nous avons décidé de moderniser la délivrance des prestations sociales et des minima sociaux, en limitant notamment les démarches administratives pour les demandeurs et en détectant